notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires mises en place depuis le mois de mars dernier. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité- je pense qu'il n'y aura pas de problème aujourd'hui ... Tous les orateurs, y compris les membres du Gouvernement, s'exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune.

en adaptant notre système de santé aux enjeux de notre temps et en permettant à chacun d'accéder à des soins correspondant à sa situation. La crise sanitaire a été une épreuve de vérité pour notre système de santé en révélant à la fois ses atouts et ses faiblesses. Depuis plusieurs années, nous le savons,

Elles sont le reflet des évolutions et des grandes mutations de notre société. La figure rassurante du médecin de famille qui prenait les décisions de santé, qui était joignable à toute heure du jour et de la nuit

et à quel point ils sont prêts à le faire encore davantage demain, en particulier dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé qui émergent et se structurent dans les territoires afin de garantir l'accès de chacun à un médecin traitant. Ce combat est fondamental, car le médecin traitant est, et doit rester, le gage d'un suivi au long cours, d'une prise en charge globale, intégrant une dimension à la fois préventive et curative et contribuant à la bonne orientation des patients dans notre système de santé.

ici, au sein de la commission, et qui, par leur contribution, proposent des solutions très concrètes pour améliorer l'accès aux soins dans notre pays. Pour éviter les situations d'engorgement des urgences, ce texte prévoit la création d'une catégorie nouvelle de structures de santé, à mi-chemin entre la médecine générale traditionnelle et les services d'urgence les points d'accueil pour soins immédiats. Cette catégorie est, sur le fond, pertinente, car nous savons que beaucoup d'admissions aux urgences ne répondent pas aux critères de la médecine d'urgence.

aux critères de la médecine d'urgence. Une signalétique spécifique, qui reste à définir, permettra d'identifier ces structures et d'orienter le patient vers celles-ci, contre le réflexe, puisque c'est bien devenu un réflexe, d'aller aux urgences. La gradation des soins ne doit pas être une notion technique, voire abstraite, pour nos concitoyens ; elle doit être une réalité de terrain. De ce point de vue, cette proposition de loi est un outil très concret pour apporter une réponse juste, pertinente, aux soins requis. requis. Il faut bien le dire, entre la consultation chez son médecin traitant et l'admission dans un service d'urgence, il y a toute une série de nuances, des degrés de gravité divers. On peut avoir besoin de soins immédiats sans pour autant requérir l'intervention de la médecine d'urgence. Autrement dit, l'ambition de cette proposition de loi est non pas de créer une couche supplémentaire,

sur la bonne coordination des collectifs de soins, sur les territoires. C'est l'un des grands enjeux de la concertation qui a été lancée par le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran. La crise sanitaire que nous traversons a conduit chaque service à se réinventer,

nous ont rappelé avec force une évidence simple : la santé est au coeur des priorités de nos concitoyens. Au moment où s'engage le Ségur de la santé, la proposition de loi du député Cyrille Isaac-Sibille dont nous allons débattre n'a pas l'ambition de refonder notre système de soins. Elle apporte une réponse ponctuelle, mais néanmoins concrète et pragmatique, à des réalités que nous sommes nombreux à constater. Ces réalités, ce sont les angoisses de nombre de nos concitoyens dans les territoires où la démographie médicale est fragile Ces réalités, ce sont aussi les difficultés, en partie corrélées, résultant de l'engorgement des services d'urgence, dont la fréquentation a plus que doublé en vingt ans,

En effet, les services d'urgence assurent une prise en charge complète, en un seul lieu et sans avance de frais. Ils offrent une réponse à une urgence médicale ressentie, que les patients ne trouvent pas toujours, dans les mêmes conditions, auprès des professionnels de ville.

Les points d'accueil pour soins immédiats (PASI), instaurés par la proposition de loi visent à assurer, pour des soins qui ne relèvent pas de l'urgence médicale, comme la petite traumatologie, une prise en charge intermédiaire entre le cabinet médical et le service d'urgence. Cette offre de soins graduée serait dimensionnée aux besoins médicaux des patients, avec un accès direct, ou organisé, à des plateaux techniques,

Elle présenterait les mêmes garanties d'accès financier aux soins, notamment par l'application du tiers payant. Toutes les auditions l'ont démontré, c'est là une exigence de chacun. Elle serait enfin aisément identifiable par une signalétique spécifique : par exemple une croix orange, comme le propose l'auteur du texte, en référence à la croix rouge des urgences et à la croix verte des pharmacies. L'instauration du label « PASI » permettra de rendre visibles et lisibles des structures qui existent pour certaines d'ores et déjà, au sein d'une maison, d'un centre de santé ou adossées à un hôpital de proximité. Les PASI s'inspirent en effet d'expériences de terrain diverses, résultant parfois de la transformation de services d'urgence surdimensionnés, parfois de l'initiative de professionnels libéraux. ont vocation à former une « réponse ambulatoire » à la prise en charge des soins non programmés, en complémentarité de Ma santé 2022 ou du pacte de refondation des urgences et des mesures progressivement mises en place pour accompagner la structuration des acteurs de la médecine de ville et le déploiement de l'exercice coordonné. En ce sens, les évolutions apportées au texte par l'Assemblée nationale ont permis d'articuler les PASI avec les projets de territoire en cours de formalisation, notamment ceux qui sont portés par les professionnels de santé dans les CPTS, comme l'a rappelé M. le secrétaire Si l'initiative est bienvenue, j'entends également certaines réserves que ce texte peut susciter ; nos débats en commission s'en sont fait l'écho. Ces réserves sont autant de points de vigilance auxquels il nous faudra être attentifs afin d'emporter l'adhésion des professionnels de santé. Un premier écueil serait de promouvoir une approche consumériste du soin. Nous aurons, lors de l'examen des amendements, un débat sur la notion de « soins immédiats », qui peut, à certains égards, induire cette perception. Au-delà des questions de vocabulaire, l'enjeu de la régulation sera déterminant pour assurer la pertinence des prises en charge et éviter tout appel d'air. Cette régulation médicale devra être cohérente avec les initiatives des professionnels dans les territoires ou avec le projet de numéro unique- le service d'accès aux soins envisagé par le Gouvernement. En outre, l'information des patients sur l'offre de soins disponible, laquelle est à ce jour largement insuffisante, sera un corollaire afin d'éviter tout risque de confusion en cas d'introduction dans le paysage sanitaire d'une croix orange. Un second écueil serait de déstabiliser l'organisation mise en place dans les territoires en ajoutant un étage au millefeuille- cela a été rappelé en commission -, une structure en plus, déconnectée des autres acteurs, comme le craignent des syndicats de médecins. Les médecins généralistes sont les premiers acteurs des soins non programmés, et il n'est nullement question de leur dérober ce rôle. les PASI ont vocation à venir en appui de ces professionnels dans leur mission. Pour cela, l'inscription des PASI dans un projet territorial est évidemment un élément fondamental. Les ajustements que nous avons introduits dans le texte de la commission, sur ma proposition, ont eu précisément pour objectif de souligner la nécessaire complémentarité des PASI avec l'offre présente à l'échelon d'un territoire. Tout effet de concurrence serait délétère, sachant combien la ressource médicale est rare. Nous avons également tenu à mettre en avant la nécessaire articulation avec le parcours de soins coordonné, de même que l'initiative première des acteurs de santé dans la démarche de labellisation. Ce type de projet ne saurait résulter d'une approche dogmatique des agences régionales de santé.

Au final, ce texte ne résoudra pas d'un coup de baguette magique les difficultés d'accès aux soins. Il ne se substitue pas non plus aux réformes attendues de notre système de santé pour mieux répondre aux besoins. Je pense, Je pense, par exemple, aux réflexions qui doivent encore progresser sur la coopération entre les professions de santé ou sur la revalorisation des visites à domicile. Cette proposition de loi offre néanmoins un outil pragmatique et complémentaire dont les professionnels de santé pourront se saisir dans les projets de territoire en cours de formalisation. Le cadre général posé par ce texte offre, selon moi, la plasticité nécessaire pour adapter les PASI aux réalités locales, tant dans les zones urbaines que dans C'est une condition qui me semble essentielle : le cahier des charges national devra rester simple et souple pour s'adapter à cette diversité et éviter tout carcan inutile.

Il nous semble cependant qu'il est conforme à des principes que nous avons à coeur de défendre dans cet hémicycle lorsque nous débattons de l'organisation de la santé : le volontariat des acteurs de terrain, la souplesse d'adaptation aux réalités des territoires, la prise en compte des besoins des patients.

novembre 2019, alors que de nombreux services d'urgence des hôpitaux publics connaissaient depuis des mois un mouvement social. Nos collègues Laurence Cohen René-Paul Savary ont parfaitement analysé les difficultés des services d'urgence. Ils doivent être regardés non comme un point d'entrée défaillant dans le système de soins, mais comme un miroir grossissant des dysfonctionnements de l'ensemble de notre système de santé. Leurs difficultés résultent moins de leur organisation propre que de leur positionnement original au confluent, en amont, des carences de la médecine de ville et de la permanence de soins ambulatoires et, en aval, des rigidités hospitalières. Nous avons régulièrement eu l'occasion d'évoquer dans cet hémicycle et au sein de la commission des affaires sociales le problème que pose pour notre système de santé la gestion de la permanence des soins et, plus généralement, de l'accueil des soins non programmés- programmés- madame la rapporteure, je préfère cette terminologie à celle de soins immédiats, qui semble accréditer l'idée d'immédiateté. Nous avons été conduits à examiner plusieurs dispositions sur ce sujet ces dernières années avec la mise en place

je le rappelle, ont pour mission de permettre aux patients du territoire concerné d'obtenir un rendez-vous le jour même ou dans les vingt-quatre heures, dès lors qu'il s'agit d'une urgence non vitale. Depuis la signature en juin dernier de l'accord conventionnel interprofessionnel, les CPTS s'organisent sur l'initiative des professionnels de santé des territoires pour construire une offre de soins coordonnée. Le ministère de la santé estimait qu'il serait nécessaire de créer environ un millier de CPTS pour couvrir l'ensemble du territoire conformément aux objectifs du plan Ma santé 2022. Monsieur le secrétaire d'État, j'ai une première question : pouvez-vous nous donner un état des lieux de la mise en place de ces CPTS ? Par ailleurs, le pacte de refondation des urgences, annoncé en octobre dernier par Mme la ministre de la santé, prévoyait la création d'un service d'accès aux soins

Même si toutes ces initiatives ne sont pas suffisantes au regard de l'engorgement des services d'urgence, la réponse à la question qui nous est posée réside-t-elle dans la création d'un nouveau label par l'ARS ? Honnêtement, je ne le pense pas. Comme je l'ai décrit à l'instant, les points d'accueil pour soins non programmés existent déjà, mais sous d'autres appellations. Ajouter une énième structure dans l'organisation des soins ne nous semble pas pertinent, d'autant plus que le Gouvernement vient d'installer le Ségur de la santé- Mme la rapporteure l'a rappelé -, qui, je l'espère, ne sera pas que le Ségur de l'hôpital Pour conclure, monsieur le secrétaire d'État, permettez-moi de former le voeu que ce Ségur ne soit pas un catalogue de demandes, mais qu'il apporte des solutions concrètes pour améliorer les conditions de travail de tous les professionnels de santé : médecins, infirmiers, paramédicaux Je prendrai un exemple : la question du temps que les personnels, tous secteurs confondus, consacrent à leurs tâches administratives. Des solutions pratiques et rapides pour augmenter le temps médical doivent être mises en place ; tout le monde y gagnera, patients comme soignants. Monsieur le

à plus de 20 millions aujourd'hui, soit près de 30 000 personnes chaque année par structure. Les établissements publics sont en première ligne, puisque seuls 18 % de ces passages sont pris en charge par le secteur privé. Afin de désengorger les urgences hospitalières des prises en charge de patients dont le pronostic vital n'est pas engagé, ce texte crée des points d'accueil pour soins immédiats (PASI), initiative développée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces PASI seraient labellisés par les agences régionales de santé.

L'amont, l'aval, le milieu, la ville, l'hôpital, les cliniques, les obligations, les incitations, les organisations, les désorganisations, les fermetures, les rémunérations, les dotations, les abandons

les personnels se sont épuisés, lassés du manque de moyens, et les usagers des urgences se sont parfois révoltés. L'heure des décisions ne peut plus être retardée. Une crise sanitaire violente vient de nous frapper.

La réponse de notre système à un virus qui nécessitait pour une large part des soins immédiats sans gravité aura particulièrement mis en lumière le défaut de sollicitation d'une chaîne de soins associant et mobilisant l'ensemble des acteurs.

En 2020, on ne meurt plus de la canicule dans nos Ehpad ; on y meurt d'un virus et d'un défaut de soins. Alors, oui, bien sûr, réorganiser nos soins d'urgence non vitale, nos soins non programmés ou immédiats, est indispensable, impératif ! L'heure des décisions ne peut plus, ni moralement ni politiquement, être retardée. Il est des débats qui, à l'heure du post-Covid, acquièrent une acuité que beaucoup ne percevaient pas, mais qui s'impose aujourd'hui. Nous y sommes Ce texte, que l'Assemblée nationale a adopté en novembre 2019, était alors un tout petit pas. Je ne sais pas s'il était efficient, mais, en juin 2020, après cette crise, cette crise, quelle peut être la signification de la création d'un nouveau nom et d'un label par les ARS ? Jusqu'à aujourd'hui, les ARS agréaient ; maintenant, elles labellisent les législateurs que nous sommes peuvent-ils porter une réponse aussi faible à l'occasion de notre premier débat post-Covid relatif à l'organisation du système de soins ?

! Même si ses conditions d'organisation nous interpellent, même si les refus déjà exprimés par le Premier ministre, comme celui de modifier la gouvernance de nos hôpitaux- quelle erreur ! ne portent pas à l'optimisme sur ses résultats, il est prématuré et trop peu signifiant d'adopter, avant ses conclusions, une proposition de loi dont le caractère beaucoup trop trop partiel pourrait être perçu par les professionnels concernés comme une désinvolture politique. Il y a parfois loin d'une intention tout à fait louable à une action utile. Cette proposition de loi l'illustre parfaitement.

trouver. À peine un an après le vote de la loi Ma santé 2022 et alors que le Ségur de la santé se met tout juste en place, cette proposition de loi revêt pour certains un caractère presque anachronique. Nous sommes en effet nombreux à nous interroger sur le de cette proposition et sur son articulation avec les nouvelles organisations de soins. Toutefois, ayant pris connaissance de l'avis de notre rapporteure, ainsi que du vote unanime de l'Assemblée nationale, j'ai entrepris de sonder les professionnels de mon territoire afin de confirmer ou d'infirmer ce premier avis. Je dois dire que les retours ont été plutôt unanimes. Sur le fond, les objectifs sont partagés : désengorger les urgences et offrir aux patients une plus grande lisibilité sur les possibilités d'accès à des soins immédiats. Néanmoins, certains éléments nous empêchent d'y voir une véritable plus-value. La raison principale réside dans l'organisation actuelle du système de soins. Si ce système est bien évidemment perfectible, nous devons reconnaître les efforts des professionnels de santé de ville pour s'adapter, dans un contexte difficile, aux réformes successives de ces dernières années, aux nouvelles organisations et aux nouveaux acronymes : PTS, PTA, CPTS, MSP, ESP ... Je pense particulièrement aux maisons de santé pluriprofessionnelles et aux communautés professionnelles territoriales de santé, dont l'une des missions premières est bien l'amélioration de l'accès aux soins en ville, notamment aux soins non programmés. que dire aux médecins qui se sont déjà organisés sur le terrain, et qui continuent de le faire, pour garantir un accès rapide à la médecine de ville pour tous ? Que nous créons un nouveau dispositif, un énième cahier des charges et de nouvelles exigences ? ? des relations qu'ils ont nouées depuis des années avec leurs partenaires, comme SOS Médecins ou les plateaux techniques de leur territoire ? Pour ma part, je suis convaincue qu'il est préférable de consolider l'existant, en confiant pleinement aux acteurs de terrain la responsabilité de mettre en place l'organisation nécessaire pour répondre aux soins dits immédiats, comme ils le font déjà sur de nombreux territoires. L'objectif doit surtout être de clarifier le rôle de chacun auprès des services de régulation et des patients pour orienter ceux-ci correctement, en allouant à ces structures des budgets supplémentaires et en incitant davantage les jeunes médecins à s'installer en zones sous-dotées.

selon une récente communication, son taux d'application stagnerait encore à 30 % ; nous en attendons une mise en application pleine, entière et plus rapide. Par ailleurs, des inquiétudes ont émergé quant au risque d'augmenter le recours aux soins, en labellisant des points d'accueil pour soins immédiats. Ces termes pourraient laisser entrevoir une forme de self-service de la santé dans une société où l'on demande toujours plus et toujours plus vite. En outre, on crée un intervenant supplémentaire et on risque de déroger au parcours de soins, dans lequel le médecin traitant joue un rôle central. Depuis le début de la crise sanitaire, notamment pendant la période de confinement, nous avons assisté à une baisse significative du nombre de passages aux urgences et dans les cabinets médicaux. Si ces chiffres ont pu alerter sur de possibles dégradations de la santé des Français par un moindre recours aux soins, il confirme l'existence de passages inappropriés, notamment aux urgences- la Cour des comptes les a estimés à environ 3,6 millions pour la seule année 2017. pourquoi je suis convaincue que nous devrions plutôt profiter de cette période et des comportements adoptés pendant la crise pour aider les patients à mieux utiliser notre système de santé. Enfin, des incertitudes demeurent sur la question des moyens. proposition de loi entrevoit, grâce à ces PASI, une baisse des dépenses de santé, certains d'entre nous, élus ou professionnels de santé, n'en sont pas convaincus. Au contraire, l'existence de telles structures pourrait conduire à une dilution des moyens existants, notamment humains, déjà très contraints. En effet, le manque de généralistes est criant dans certains territoires, et je crains que cette proposition de loi ne vienne porter un nouveau coup à la médecine de proximité, en polarisant les soins de premier recours autour des centres d'urgence de ville, que l'on imagine plus aisément s'installer en agglomération qu'en zone rurale. Pour conclure, je dirai que tout le monde s'accorde sur les objectifs je souscris aux amendements de la rapporteure Élisabeth Doineau adoptés en commission, qui renforcent la cohérence des PASI avec l'offre de soins et le parcours santé et tentent de réaffirmer l'initiative première des acteurs du territoire dans la démarche de labellisation. Pour autant, je ne suis pas totalement convaincue qu'un nouvel outil réponde aux problématiques soulevées, en particulier dans le contexte du lancement du Ségur de la santé. Là où les organisations sont en place, là où les professionnels de terrain se coordonnent, le système fonctionne bien. Il faut donc accélérer les transformations en cours. Pour cela, un travail doit être mené, notamment sur les zones dites atones, c'est-à-dire là où les élus et les professionnels ont du mal à s'organiser. Une piste que vous pourriez reprendre pour le Ségur de la santé est de renforcer sur les territoires en difficulté une véritable ingénierie de projet. Je terminerai en rappelant que la période que nous venons de vivre a consacré la pratique de la télémédecine comme alliée indispensable de notre système de santé. C'est avec ces outils, déjà existants, et non avec des échelons supplémentaires, que nous devons penser la santé de demain.

tout d'abord, je veux associer mon groupe à l'hommage rendu aux soignants durant la crise que nous connaissons encore aujourd'hui. Bernard Jomier, depuis vingt ans, le nombre de passages aux urgences ne fait qu'augmenter dans notre pays. Il a même doublé depuis 1996. Confrontés à la douleur et à l'angoisse, nos concitoyens privilégient massivement les services d'urgence afin d'obtenir une réponse rapide et un diagnostic précis. Ainsi, en 2016, on comptait plus de 21 millions de passages aux urgences, contre 10,1 millions en 1996. Plusieurs facteurs expliquent ce recours aux urgences. Nous avons en tête l'image de services d'urgence engorgés, de personnels à bout de force, mais aussi déterminés et qui ont tenu bon.

Dans son rapport de 2017, la Cour des comptes estimait à 3,6 millions par an le nombre de passages dits « inutiles » aux urgences. Ce chiffre doit malgré tout être relativisé, puisque, selon une autre étude parue en octobre 2019, ces visites inadéquates ou inutiles seraient notamment liées à un manque patent de médecins généralistes dans nos territoires. Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des solidarités et de la santé, près de 60 % des patients se rendent aux urgences parce que les soins y sont accessibles et qu'ils peuvent y réaliser rapidement des examens complémentaires. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permet en partie de répondre à la demande croissante de diagnostic et de soins rapides des patients, par la création de points d'accueil pour soins immédiats. Ces points d'accueil auraient trois missions : assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale, lorsque le pronostic vital du patient n'est pas engagé ; caractériser l'état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu par un médecin généraliste ; orienter si nécessaire le patient vers un service d'urgence ou un service spécialisé. La crise que traversent les services d'urgence ne date pas d'hier. Elle est le fruit du manque d'investissements qui, depuis de nombreuses années, a fragilisé le secteur et impacté les conditions de travail des professionnels de santé. Nous saluons les objectifs de cette proposition de loi. Celle-ci vise à participer à une meilleure gradation de la réponse à la demande de soins non programmés, en maillant plus finement le territoire. la création des points d'accueil pour soins immédiats dédiés à la prise en charge de soins rapides des patients dont le pronostic vital n'est pas engagé constituerait un début de réponse face à l'engorgement des services d'urgence. En 2017, un rapport d'information de nos collègues Laurence Cohen, Catherine Génisson et René-Paul Savary faisait déjà état d'un changement de mentalité de la part de nos concitoyens et d'une évolution sociétale valorisant l'immédiateté de l'accès aux soins, ce qui expliquerait notamment le recours aux urgences hospitalières chez les patients. Une autre recommandation est la prévention. Celle-ci se traduit tout d'abord par une meilleure information de la population. Elle constitue l'un des enjeux importants du désengorgement des services d'urgence, auxquels on recourt parfois par méconnaissance de l'état de santé des patients. L'éducation à la santé de la population, c'est aussi permettre à chacun de savoir vers quel professionnel se tourner en fonction de son état de santé. Il nous paraît essentiel de permettre à ces points d'accueil pour soins immédiats de jouer ce rôle. Tel est l'objet de l'amendement que nous avons déposé sur ce texte.

efficaces et, surtout, les difficultés auxquelles font face celles et ceux qui, chaque jour, sauvent des vies dans des conditions toujours plus difficiles. Conscient de cette réalité- nous le sommes tous -, le Gouvernement a lancé, la semaine dernière, le Ségur de la santé. concertation avec l'ensemble des acteurs du système de santé, de l'hôpital, de la ville et du secteur médico-social fait suite à l'engagement pris par le Président de la République le 25 mars dernier dans le discours qu'il dans lequel il a exprimé son souhait qu'un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble de carrières soit conduit à l'issue de la crise. L'une des priorités est la mise en place d'organisations plus proches des territoires et plus collectives entre l'hôpital, la médecine de ville et le secteur médico-social. évidemment, l'adoption de cette proposition de loi ne sera qu'une petite pierre à l'édifice qu'il nous faut construire. Le Ségur de la santé permettra- nous l'espérons sincèrement -de refonder notre système de santé face aux difficultés rencontrées par les professionnels et les patients.

: l'organisation de notre système de santé est en pleine ébullition. La crise née de la pandémie du Covid-19 a été le révélateur des maux dénoncés depuis des années à l'hôpital. Ce texte, qui part d'un bon sentiment, ne prend pas en compte l'ampleur des difficultés et reste assez flou, puisque nous n'avons aucun élément sur le futur cahier des charges, qui sera défini

des maladies chroniques. En réalité, c'est toute la chaîne des soins qu'il faut revoir, en travaillant en profondeur sur la complémentarité entre médecine de ville et hôpital, et non sur la mise en concurrence du public et du privé. Si les cliniques privées ont été si peu mises à contribution durant la crise du Covid-19 pour soigner les malades, c'est en partie le résultat des politiques de tarification à l'activité et de cette mise en concurrence, qui les ont conduites à se spécialiser dans les soins rentables à fort remboursement. Le risque n'est-il pas que cette proposition de loi permette aux cliniques commerciales de prendre en charge les patients qui en ont les moyens ?

pratiquant le tiers payant, ce que nous défendons totalement, elle ouvre la porte aux structures pratiquant des dépassements d'honoraires, sous réserve simplement que le patient l'idée d'encourager les médecins libéraux à s'organiser sur leur territoire est tout à fait juste, ce texte méconnaît les réalités. Dans mon département du Val-de-Marne, il existe douze structures, dénommées « SAMI », qui assurent les urgences médicales le soir, le week-end et les jours fériés. Ce système fonctionne grâce, d'une part, à l'implication du conseil de l'ordre départemental des médecins ainsi que d'une équipe de médecins volontaires et, d'autre part, à l'engagement de collectivités, qui participent à certains frais. Mais, aujourd'hui, ces médecins volontaires ont vieilli et ne trouvent pas de relève. Le fait que les SAMI soient labellisés PASI ne changera rien à l'affaire. Il serait d'ailleurs peut-être temps, monsieur le secrétaire d'État, de revenir sur le décret qui a supprimé les gardes des médecins le soir et le week-end. Ah oui ! Sachant votre qualité d'écoute, je compte sur vous pour faire remonter ce voeu à M. le ministre des solidarités et de la santé. Cette proposition de loi cherche à trouver une solution, en distinguant les soins urgents des soins immédiats, qui n'entraîneraient pas de risque pour la survie des patientes et des patients. Pour y parvenir, elle propose d'associer plus fortement les professionnels de santé de proximité autour d'un plateau technique et au sein d'une CPTS, ce qui concerne notamment les maisons de santé et les centres de santé.

En fait, les différents plans qui se sont succédé, notamment lors du passage de Mme Buzyn au ministère, n'ont pas rompu avec la logique de restrictions budgétaires qui plombe notre système de santé. Le plan Ma santé 2022 met notamment à mal les hôpitaux de proximité, en remettant en cause leurs missions,

particulièrement mobilisés depuis plus d'un an et des enseignements de la pandémie du Covid-19, le Gouvernement va-t-il enfin remettre à plat l'intégralité de notre système de soins ? Les solutions passent, en plus de ce que j'ai énoncé, par l'augmentation globale du budget de l'hôpital- vous savez que nous avons des propositions de nouveaux financements pour y parvenir -, l'ouverture de lits d'amont et d'aval des urgences et la revalorisation des professionnels de santé et du médico-social, avec une augmentation de leurs salaires et une progression de leur statut. Il ne suffit pas de dire, dans cet hémicycle, que l'on soutient

Parce que nous ne pouvons ignorer la gravité de la crise de notre système de santé, nous ne pouvons nous contenter d'un sparadrap sur une jambe de bois. C'est pourquoi notre groupe votera contre ce texte. La parole

La proposition de loi du député Cyrille Isaac-Sibille vise à créer des points d'accueil pour soins immédiats sur l'ensemble du territoire, avec pour objectifs d'améliorer l'accès aux soins et de désengorger les urgences. Je souhaite saluer son travail ainsi que celui de notre rapporteure, Mme Élisabeth Doineau. Le développement de ces pôles est une mesure de bon sens. Nos services d'urgence prennent en charge une part significative de soins non programmés n'entrant pas du tout dans le champ de leurs missions.

La présente proposition de loi vise à mettre en place une solution avec des points d'accueil pour soins immédiats (PASI) sur tout le territoire, les patients y étant orientés

« point d'accueil pour soins non programmés », car le terme « immédiat » peut évoquer, d'emblée, une urgence, laquelle est traitée par le SAMU et le service d'urgence. Le PASI a été envisagé, dans un premier temps, au sein des établissements de santé, mais les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)

Les structures d'urgence accueillent aujourd'hui, en moyenne, plus de 30 000 patients par an. Cette situation met en évidence l'importance de la demande de soins non programmés dans notre pays et le déséquilibre de notre organisation. Cette demande est alimentée par divers facteurs, que nous connaissons tous : le vieillissement de la population, l'exigence croissante, de la part des patients, d'un diagnostic et d'une prise en charge la désertification médicale et la mauvaise répartition des généralistes sur notre territoire national. J'y ajouterai la décision de revenir sur la permanence des soins, qui a été prise voilà maintenant quelques années. Les données recueillies par la Drees dans son enquête nationale de 2013 sont, de ce point de vue, alarmantes. Ainsi, un cinquième des patients se rend aux urgences par défaut.

Plus grave encore, près des deux tiers des patients qui se rendent aux urgences y vont pour des raisons tenant à l'accessibilité des soins. Les patients se dirigent vers les services d'urgence alors même qu'ils savent qu'ils vont probablement devoir attendre plusieurs heures avant d'être examinés- Les services d'urgence assurent une part importante des soins non programmés, qui ne relèvent pas de leurs missions et pourraient être pris en charge par d'autres structures. L'impossibilité de trouver une réponse en médecine de ville impacte fortement le recours aux urgences.

Une médecine de ville mieux organisée et dotée de bons outils devrait normalement pouvoir accueillir une proportion plus importante de ces patients. La situation est grave, pour plusieurs raisons. Elle crée une surcharge d'activité des services d'urgence, qui sont aujourd'hui au bord de l'implosion et engorgés, faute d'alternative. Elle crée aussi un surcoût important pour l'assurance maladie. À plusieurs reprises, nous avons tenté de résoudre cet embouteillage des services d'urgence, que nous connaissons tous sur nos territoires. Nous avons créé des centres de santé, des maisons de santé, des maisons médicales de garde, des hôpitaux de proximité. Pour autant, les bénéfices de ces dispositifs restent en deçà des attentes. Ils apportent une réponse encore insuffisante et disparate sur le territoire. Surtout, les différences statutaires entre les diverses organisations

CPTS, nous répondrions à une forte demande de nombreux patients qui fréquentent les services d'urgence. Or, à ce jour, il est difficile pour des médecins libéraux de disposer du matériel leur permettant d'effectuer des soins de première urgence. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire

cela soit lisible pour la population : le citoyen doit être en mesure d'identifier une gradation dans l'offre de soins, du soin non programmé à l'urgence vitale. Tel est l'objet de cette proposition de loi, dont l'ambition est de contribuer à apporter une réponse rapide aux besoins de nos concitoyens, en labellisant et en rendant identifiables, pour les patients, des structures qui existent d'ores et déjà. La reconnaissance des PASI permettra de mailler le territoire d'une offre de soins non programmés graduée.

Les PASI permettront aux patients de mieux comprendre la réponse de l'offre de soins compte tenu de leur état de santé. Ils permettront de désengorger les services d'urgence, comme je l'ai évoqué au début de mon intervention. Ils offriront un choix supplémentaire au médecin régulateur du SAMU, qui pourra décider d'orienter soit vers un PASI, soit vers un service d'urgence, ce qui accroîtra notre maillage territorial sans créer de nouvelles structures. Le PASI sera un label qui pourra être obtenu par les différentes structures de soins. Il ne sera pas imposé par l'administration. Il ne sera obtenu que sur l'initiative des professionnels de santé et coordonné sur un même territoire par les CPTS, pour éviter les phénomènes de concurrence. Les structures ainsi labellisées seront complémentaires de l'offre des hôpitaux de proximité et de celle de la médecine de ville classique.

Il s'agit d'un texte d'opportunité, visant à répondre à la situation dramatique dans laquelle se trouvent les urgences hospitalières, dont les personnels dénoncent régulièrement leurs mauvaises conditions de travail, le manque de considération, l'épuisement physique, le manque de lits ou encore les conditions déplorables d'accueil des patients.

L'acte médical est devenu, aujourd'hui, un bien de consommation courant. Or la médecine de ville ne répond pas aux critères d'exigence de certains patients, au premier rang desquels figure la possibilité d'être reçu immédiatement en cabinet pour connaître précisément son état de santé ou recevoir des soins primaires. Les services d'urgence des hôpitaux sont devenus le lieu vers lequel tout un chacun se tourne. On en connaît les conséquences humaines, matérielles et financières, car, au malaise profond des personnels soignants, lié à la surcharge d'activité, il faut ajouter les surcoûts considérables pour l'assurance maladie. Cette proposition de loi a-t-elle les moyens de ses ambitions ? L'intention est louable : désengorger les services d'urgence des hôpitaux, en créant des points d'accueil pour soins immédiats pouvant réaliser des soins non programmés dès lors que le diagnostic vital du patient n'est pas engagé. Dans les faits, ce texte ne révolutionnera pas l'organisation du système de santé, tant s'en faut. Il est déposé moins d'un an après l'entrée en vigueur de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, dont l'objet, il faut le rappeler, était de décloisonner toutes les parties prenantes- médecine de ville, hôpitaux, secteurs médico-sociaux -et de tendre vers un exercice plus ouvert, pluriprofessionnel et coordonné. Nous l'examinons alors que le Président de la République vient d'annoncer le Ségur de la santé, censé identifier les maux qui affectent notre système de santé Pis, au lieu d'apporter de la souplesse dans l'organisation des soins, cette proposition de loi procède d'une vision technocratique, en donnant aux agences régionales de santé compétence, d'une part, pour labelliser et rendre identifiables par les patients des structures qui existent déjà et, d'autre part, pour délivrer des habilitations. De telles initiatives sont, de mon point de vue, vouées à l'échec tant que l'on ne traitera pas le problème de base, à savoir l'accès aux soins sur tout le territoire. Je pense en particulier au monde rural et aux territoires de montagne, mais également à la question de l'inégale répartition des professionnels de santé et à celle de la démographie médicale, qui sont fondamentales. À quoi bon créer des structures, si l'on ne dispose pas de personnel pour les faire vivre ? J'attends plutôt du Gouvernement qu'il laisse les professionnels s'organiser localement et qu'ils privilégient les initiatives émergeant partout en France pour rendre les soins accessibles au plus grand nombre. Ces projets sont la plupart du temps portés par des élus ou par des communautés de soignants qui souhaitent être utiles et exercer différemment leurs compétences, au service de l'intérêt collectif. J'en veux pour preuve une offre innovante qui a vu le jour récemment à Moigny-sur-École, village de 1 200 habitants de mon département de l'Essonne. Le premier centre de télémédecine d'Île-de-France y a ouvert ses portes au début de l'année 2019, au coeur d'un territoire- le Gâtinais français -marqué par le vieillissement de sa population et la perspective du départ à la retraite, d'ici à cinq ans, de 50 % des médecins y exerçant. L'objectif de la municipalité était de faciliter l'accès aux soins des patients, de telle sorte qu'il n'y ait pas de rupture de suivi ou de prescription. L'autre volet du projet était de libérer du temps de soins pour les médecins généralistes du territoire, par des téléconsultations performantes, centrées sur l'expertise médicale, le diagnostic et la prescription. L'expérimentation de la télémédecine en zone rurale fait d'ailleurs partie des actions développées dans le plan Santé 2019-2023 du département de l'Essonne pour lutter contre la désertification médicale et désengorger les urgences hospitalières. Je ne peux conclure mon propos sans évoquer la maison de santé hors les murs de Verrières-le-Buisson, fruit d'une collaboration exemplaire entre la municipalité et des professionnels de santé. Monsieur le secrétaire d'État, faites confiance aux territoires pour créer et innover dans plutôt que d'imposer des solutions toutes faites et bien peu efficaces comme celle que comporte cette proposition de loi ! C'est à cette condition que notre système de santé retrouvera sa crédibilité et sa capacité à soigner nos concitoyens, où qu'ils résident et quelles que soient leurs pathologies, légères ou graves. Pour les raisons que j'ai exposées, le groupe Les Républicains ne votera pas ce texte. La parole

pris part aux réponses qui s'organisaient sur les territoires face à la crise dans laquelle nous nous trouvons encore. En ce qui concerne le SAS, la crise a apporté des enseignements importants,

dans un certain nombre de structures, reçoivent déjà sans rendez-vous des patients dont l'état nécessite des soins immédiats sans urgence vitale. La volonté première de ce texte est de participer au désengorgement des services d'urgence des hôpitaux, ce qui nécessite également d'aborder la question de la prévention et de l'éducation de la population à la santé.

Le Gouvernement est attaché à garantir que les points d'accès pour soins immédiats s'inscrivent dans des relations de coopération entre acteurs d'un même territoire, autour de l'organisation des soins non programmés. le PASI dans un projet de CPTS constitue une garantie essentielle de cette dynamique de coopération entre acteurs et de la cohérence des solutions apportées sur un même territoire.

été maintenue par la commission -, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi, dans la mesure où tous les articles qui la composent auraient été rejetés ou supprimés. Il n'y aurait donc pas d'explications de vote sur l'ensemble.

Le scrutin est ouvert.

le résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,

n'a pas adopté. Les articles de la proposition de loi ont été successivement rejetés ou supprimés par le Sénat. Je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée.

la demande du groupe Union Centriste, la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

est à Mme la secrétaire d'État. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les abus en matière de démarchage téléphonique et l'usage frauduleux des numéros surtaxés sont une nuisance pour nos concitoyens. Pour certains, c'est un supplice quasi quotidien qui se produit de manière intempestive. Pis, ces démarchages frauduleux entraînent parfois des préjudices financiers qui peuvent être très significatifs. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite lutter contre ces pratiques. Il s'agit là d'un sujet complexe, dont témoignent les nombreux débats sur cette proposition de loi. Il nous faut en effet trouver un subtil équilibre permettant d'assurer l'impérieuse protection de nos concitoyens sans pour autant pénaliser les acteurs respectueux de la loi. Je voudrais tout d'abord souligner l'importance et l'intérêt des mesures que comporte ce texte et du travail qui a été accompli. En première lecture, des dispositifs visant à renforcer significativement la protection des consommateurs ont déjà été votés le renforcement de leur information dans les contrats et lors de la prospection commerciale, une obligation plus forte pour les entreprises ayant recours au démarchage téléphonique de s'assurer qu'elles respectent bien la liste d'opposition, des sanctions alourdies pouvant aller jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale et une publication systématique de ces sanctions aux frais du professionnel, un mécanisme plus réactif et plus sécurisé juridiquement de suspension et résiliation des numéros surtaxés des opérateurs indélicats, avec une faculté de saisine du juge des référés par la DGCCRF.

Ont notamment été mis en place un encadrement plus strict des conditions de mise en oeuvre du démarchage téléphonique, notamment des jours et des heures auxquels il peut être pratiqué, une responsabilisation accrue des professionnels, avec présomption de responsabilité du professionnel ayant tiré profit des sollicitations commerciales, un meilleur encadrement des exceptions à la liste d'opposition dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. Les travaux menés en commission par votre assemblée sont également venus consacrer ces évolutions dans un souci d'amélioration du texte. Je voudrais cependant revenir sur la mesure d'interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, qui a été supprimée en commission. Cette interdiction, je le redis, est demandée par les associations de protection des consommateurs.

À l'heure où nous devons faire de la transition environnementale une priorité pour l'avenir de notre pays, nos concitoyens doivent pouvoir avoir confiance dans la rénovation énergétique. Je le rappelle, le plan de lutte contre la fraude dans le secteur de la rénovation énergétique, que j'ai lancé conjointement avec le ministre du logement et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire le 12 novembre dernier, comporte divers volets, dont une campagne de sensibilisation du grand public, qui a été déployée à l'automne dernier, et des actions pour mieux protéger les consommateurs, qui font l'objet de travaux au Conseil national de la consommation. Si nous voulons que ce plan de lutte soit efficace et cohérent, nous recommandons de voter une interdiction du démarchage dans ce domaine particulier. Une telle interdiction se justifie, je le répète, par le nombre anormalement anormalement élevé de problèmes liés à ce type de démarchage, par le fait qu'il aboutit, en règle générale, à des fraudes et par la visibilité des accompagnements financiers que vous avez votés en matière de rénovation thermique. Le démarchage postal et par courriel reste permis, ainsi que la possibilité de se faire référencer par des sites de confiance. Les possibilités des experts de ces métiers pour faire connaître leurs offres sont donc nombreuses. Pour autant, nous avons entendu les craintes au sujet d'une mesure d'interdiction trop large et susceptible de perturber des professionnels qui ont des métiers connexes et ne font pas de la rénovation thermique leur activité principale. C'est pourquoi il vous est proposé de maintenir, dans certains cas, la faculté pour les professionnels de proposer à un client de réaliser des travaux. Le Gouvernement a ainsi déposé un sous-amendement visant à introduire la possibilité pour un professionnel de réaliser la prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique, compte tenu de l'antériorité et de la nature de la relation contractuelle entre le professionnel et ses clients, ainsi que de la proportion d'aides publiques liées à la rénovation énergétique dans le chiffre d'affaires du professionnel dans des conditions fixées par décret. Au total, la mesure d'interdiction soumise à votre vote est proportionnée et s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de lutte contre la fraude dans le secteur de la rénovation énergétique porté par le Gouvernement. Celui-ci permettra de renforcer la protection des consommateurs et de mettre fin aux sollicitations indésirables.

C'est la raison pour laquelle je propose d'encadrer par voie réglementaire les jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques sont autorisées et de ne pas inclure dans cet encadrement la fréquence des appels, eu égard à la grande diversité des secteurs d'activité, ainsi que des produits et services concernés. Nous souhaitons également maintenir le principe d'une responsabilité de plein droit du professionnel ayant tiré avantage d'un démarchage téléphonique illicite. Il convient non seulement que le professionnel ne soit pas à l'origine de la violation des règles d'opposition au démarchage téléphonique pour échapper à la mise en cause de sa responsabilité,

sur la lutte contre l'usurpation de numéros nationaux dans le cadre d'appels internationaux et l'authentification des appels. Il est dommage pour les citoyens qu'elles n'aient pas été maintenues par votre assemblée du fait de la règle de l'entonnoir, car elles leur apportent un réel bénéfice. Mesdames, Mesdames, messieurs les sénateurs, dans le cas des abus et fraudes dont il est question ici, l'ingéniosité des fraudeurs rend la tâche des services de l'État difficile. C'est pourquoi le renforcement du cadre normatif que prévoit cette proposition de loi est indispensable. Il viendra soutenir l'action de la DGCCRF et de tous les services de l'État mobilisés pour lutter contre ces fraudes. C'est en conjuguant une loi forte et efficace avec une action concrète sur le terrain que nous serons à même de répondre à l'attente de nos concitoyens : faire cesser les appels frauduleux et le démarchage téléphonique intempestif.

il en est d'ailleurs aussi le rapporteur -, après son adoption par l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier. Composée initialement de six articles, la proposition de loi en comptait onze lors de sa transmission au Sénat et quatorze lors de son adoption en première lecture le 21 février 2019-

protection du consommateur et développement de l'activité économique. Nous souhaitons parvenir à un bon équilibre à cet égard. Selon moi, nous n'en sommes pas si loin, si le Sénat, dans sa sagesse, ne démolit pas ce à quoi nous sommes parvenus.

été adopté conforme par la commission. Il redéfinit le champ de l'exception contractuelle permettant à un professionnel de contacter un consommateur inscrit sur Bloctel, en la restreignant aux sollicitations en rapport avec l'objet d'un contrat en cours, qui peuvent également porter sur des produits complémentaires- c'est une nouveauté. Cette nouvelle rédaction présente l'avantage d'être plus protectrice des consommateurs que le droit actuel,

Toujours dans le même état d'esprit constructif, la commission n'est pas revenue sur la suppression de deux articles par l'Assemblée nationale, à savoir l'article 1A concernant les modalités d'inscription à Bloctel par téléphone- il était en réalité déjà satisfait par les textes, cher monsieur Sueur

la commission n'a pas adopté l'ensemble du texte conforme, en raison de trois dispositions contestables introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Tout d'abord, nos collègues députés ont interdit, à l'article 1, le démarchage téléphonique aux professionnels qui vendent des équipements ou des travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d'économies d'énergie ou la production d'énergie renouvelable. Je vous proposerai de supprimer cette disposition- des amendements nous demanderont de la réintroduire

de se prononcer. Ensuite, l'Assemblée nationale a adopté, à l'article 6, des dispositions nouvelles, que la commission a supprimées au titre de la règle dite de l'entonnoir. Elles visaient à imposer aux opérateurs de filtrer

que, parmi les mesures que peut demander la DGCCRF au juge judiciaire en référé ou sur requête, figure la suspension de l'attribution de nouveaux numéros aux exploitants de numéros surtaxés pendant cinq ans au maximum. Une telle durée a semblé excessive à la commission, qui l'a donc ramenée à six mois. Enfin, la commission a apporté d'autres modifications moins substantielles à l'article 1 visant à clarifier le caractère réfragable de la présomption de responsabilité du professionnel qui méconnaîtrait ses obligations en matière de démarchage téléphonique et à préciser le texte sur les obligations déontologiques auxquelles les professionnels seraient désormais soumis. Dans la discussion que nous allons avoir, de nombreux amendements reviennent sur le sujet dit de l'.

À bon entendeur salut ! Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain ! Ce n'est pas parce qu'il y a trop d'abus qu'il faut refuser tous les démarchages téléphoniques et les interdire, comme certains voudraient le faire.

inscrite dans l'espace réservé au groupe Union centriste, limité à une durée de quatre heures. Dans ces conditions, je me verrai dans l'obligation de lever la séance à dix-huit heures trente-huit. Si nous n'avons pas achevé l'examen de ce texte, il appartiendra à la conférence des présidents d'inscrire la suite de cette proposition de loi à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

ont renoncé à décrocher leur téléphone. Pourquoi ? Parce que, plusieurs fois par jour, elles sont assaillies d'appels pour les démarcher pour toutes sortes de choses. Les maires de ces petits villages font valoir qu'en cas d'inondation- ce n'est pas une fiction -ou d'incendie la seule manière de prévenir les habitants est de leur téléphoner. ces personnes sont tellement écoeurées de ces abus constants qu'elles n'utilisent plus le téléphone. On ne peut donc pas les prévenir d'un danger.

mais ne disposent pas toujours de la compétence nécessaire, si bien qu'il y a des tromperies, des duperies, une utilisation fallacieuse de l'argent de l'État

de mettre fin à ce qui est devenu un véritable fléau pour nos concitoyens.

je venais d'arriver de recueillir le consentement préalable du consommateur en amont de toute activité de démarchage par voie téléphonique devrait être la règle. C'est la seule solution pour éviter les dérives constatées, qui confinent vraiment, parfois, au harcèlement et qui, en

Trop souvent, les consommateurs ignorent les droits qui leur sont reconnus dans le code de la consommation- peut-être moins, désormais, ceux qui figurent dans les textes relatifs à la protection des données personnelles, qu'il s'agisse de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du règlement général sur la protection des données, entré en vigueur en 2018. Les problèmes, dans le domaine du démarchage, sont donc parfaitement connus. Eu égard aux pratiques commerciales agressives de nombreuses sociétés de télémarketing n'hésitant pas à appeler les personnes plusieurs fois dans le même mois, à des horaires inopportuns, en soirée ou le week-end, il paraît totalement indispensable de renforcer les droits des citoyens. C'est pourquoi on ne peut que regretter la position encore très timorée de la commission, qui a édulcoré le texte. On évoque volontiers les consommateurs

échoué. L'approche plus modérée des auteurs de la présente proposition de loi devrait permettre d'aboutir à un compromis. Elle conserve le régime actuel de la désinscription tout en le rendant plus efficace. Son objet est aussi plus large et plus actuel, puisqu'il inclut la lutte contre les appels frauduleux, phénomène hélas répandu.

Appels internationaux, messages vocaux préenregistrés et publicitaires sous un faux numéro ... Selon les chiffres de l'enquête de l'UFC-Que Choisir de 2017, chaque foyer est démarché téléphoniquement 4 fois par semaine en moyenne. Ce chiffre monte à 4,4 fois par semaine pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

l'article 2, la réalisation d'un audit de la société Opposetel, délégataire du service Bloctel, afin de relever les dysfonctionnements, d'améliorer le service et d'optimiser les moyens

aux opérateurs de communications électroniques de suspendre l'accès à un numéro surtaxé affecté à un service fraudeur. Il est important de rappeler que le secteur du démarchage téléphonique emploie aujourd'hui directement plus de 56 000 personnes en France, y compris au sein de TPE et de PME de nos territoires.

mieux protéger les consommateurs et de renforcer l'efficacité des mécanismes d'opposition du service Bloctel sans pénaliser les acteurs respectueux de la loi, de mieux réguler le démarchage, de faire cesser ces nuisances et de sanctionner les fraudes sans ébranler le secteur.

d'un démarchage ou encore la création d'un régime de données ouvertes applicable à l'organisme gestionnaire du service Bloctel, afin d'en renforcer le contrôle. Il a permis, enfin, l'acceptation en commission de modifications du texte intervenues à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur des sujets essentiels qui faisaient encore l'objet d'une divergence de fond. Je pense notamment à l'article 5 relatif à l'encadrement du démarchage téléphonique en cas de relations contractuelles préexistantes. La rédaction de compromis introduite par l'Assemblée nationale et validée par notre rapporteur limite l'exception contractuelle aux clients d'un contrat en cours ou à des sollicitations en rapport avec l'objet du contrat ou portant sur des produits ou services afférents ou complémentaires.

certaines modifications introduites en commission par notre rapporteur relatives aux obligations imposées aux professionnels du démarchage téléphonique, s'agissant par exemple de la fixation de la fréquence des appels ou de la présomption de responsabilité s'appliquant aux professionnels ayant tiré profit d'un démarchage téléphonique litigieux.

et la lutte contre le démarchage subi. Car c'est bien de cela qu'il s'agit : une contrainte, pour ne pas dire une plaie, pour un grand nombre de nos concitoyens Vous vous levez le matin et allumez votre télévision ou votre radio : publicité ! Vous lisez votre journal ou surfez sur internet : publicité ! Vous vous rendez sur votre lieu de travail : publicité dans les transports et dans les rues ! Et quand vous pensez pouvoir être enfin tranquille, c'est votre téléphone qui sonne à répétition. En définitive, qui paie les conséquences de cette stratégie agressive ? en premier lieu- j'y reviendrai plus longuement en présentant l'un de nos amendements -, les salariés du secteur. Mal rémunérés, mis en concurrence, surveillés jusqu'à l'extrême et totalement déshumanisés, ils sont pris entre le marteau et l'enclume : d'un côté, les méthodes scandaleuses de leur direction ; de l'autre, les réactions parfois virulentes des personnes contactées. Ce sont, en second lieu, les citoyens.

De plus en plus se pose, dans le débat public, la question de ces « petits métiers », souvent aliénants, qui pourraient disparaître sans que la société ne vacille sur sa base. Il est certain que le démarchage téléphonique entre largement dans cette catégorie. est en effet la finalité de cette activité ? La libre information et le conseil aux clients ? Quiconque a déjà eu à répondre à l'appel d'un démarcheur sait bien que c'est faux. La préservation de l'emploi ? Il est vrai que le secteur emploie 56 000 personnes en France et rapporte plus de 2 milliards d'euros par an. Mais pour qui ? Pour quoi ? Pour quelle utilité sociale ? D'ailleurs, quitte à parler d'emplois, parlons un peu de la pratique, plus répandue que dans la majorité des autres secteurs économiques, de la délocalisation et de la sous-traitance dans des pays francophones au droit du travail plus faiblement

au-devant de graves problèmes en termes de développement économique et social des pays en question. Pour faire face à cette situation, le législateur a pris des mesures. La plus emblématique d'entre elles est la création des listes d'opposition la liste rouge en 1978, puis Pacitel en 2011, enfin Bloctel en 2016. Malheureusement nous sommes restés au milieu du gué. Bloctel illustre bien, d'une certaine façon, la faiblesse organisée de la régulation du secteur. Sa première faiblesse tient à son principe même : faire reposer la régulation du démarchage sur l'initiative du consommateur conduit toujours à laisser sur le bas-côté les personnes non informées ou ne maîtrisant pas l'outil. L'accord préalable du consommateur pour tout démarchage téléphonique doit être la norme, et non l'exception. Sa seconde faiblesse est celle des moyens de contrôle et de sanction. N'oublions pas que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes voit fondre, depuis plusieurs années, ses effectifs et ses dotations. Comment expliquer autrement que plus de 200 000 personnes inscrites sur Bloctel se plaignent encore de démarchage agressif ? Comment expliquer autrement que les entreprises rechignent toujours autant à nettoyer leurs fichiers de contacts ?

croyez-vous vraiment qu'un démarcheur va prendre le temps d'informer son correspondant de ses droits et de présenter Bloctel, alors que son appel est minuté et scruté par sa hiérarchie, comme l'ont montré plusieurs enquêtes ?

Nous espérons tous que nos débats permettront d'aboutir prochainement à un texte conciliant la tranquillité des Français à leur domicile avec la possibilité, pour les professionnels, de développer leur activité. Le démarchage téléphonique abusif est devenu une véritable nuisance, et nos concitoyens sont unanimes à dénoncer les appels intempestifs reçus à leur domicile. Ce constat de départ ne doit pas nous faire oublier que le démarchage téléphonique est une pratique commerciale légale et que ce secteur représente de nombreux emplois directs en France : plus de 55 000, dont pas moins de 15 000 dans les seuls Hauts-de-France. Il nous faut prendre garde à ne pas menacer ces emplois, car les centres d'appels représentent souvent un premier accès à l'emploi pour des personnes fragiles. En outre, ces emplois sont flexibles et permettent à des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler à plein temps de percevoir un complément de revenu. Ce n'est donc pas le démarchage vertueux qu'il faut interdire, mais bien la fraude au démarchage. Les entreprises qui pratiquent le démarchage de manière illégale jettent l'opprobre sur tout le secteur : appels surtaxés illégaux, automates intempestifs, appels-pièges, usurpations de numéros : autant de pratiques frauduleuses qui excèdent nos concitoyens.

! Ne nous y trompons pas : la cible, ce sont bien les fraudeurs, et non le démarchage téléphonique en tant que tel. Sur le fond, je tiens à saluer les travaux de la commission, qui a souhaité revenir sur trois modifications opérées par l'Assemblée nationale. nationale. Nos collègues députés ont interdit le démarchage téléphonique aux professionnels qui vendent des équipements ou des travaux « destinés à des logements et permettant la réalisation d'économies d'énergie ou la production d'énergies renouvelables

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté des dispositions nouvelles, sans aucun lien avec celles qui restent en discussion, visant à imposer aux opérateurs de filtrer les appels internationaux qui utilisent frauduleusement un numéro national et de mettre en oeuvre un mécanisme d'authentification des appels.

pour qu'il suspende l'attribution de nouveaux numéros aux exploitants de services à valeur ajoutée jugés frauduleux pendant une durée maximale de cinq ans. La durée de cette mesure semble excessive s'agissant de procédures d'urgence et de décisions rendues par ordonnances à titre provisoire. Je suis heureux que la commission l'ait ramenée à six mois. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la question du démarchage téléphonique abusif ou frauduleux nous concerne tous. Ce phénomène est dénoncé partout en France. Aussi, eu égard à l'exaspération légitime de nos concitoyens face à ce démarchage excessif et peu scrupuleux, est-il de notre devoir d'agir, mais avec prudence, car tout démarchage n'est pas condamnable ! Conscient tant des enjeux relevant du respect de la vie privée et de la tranquillité

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, une fois encore, nous examinons cette proposition de loi dont l'examen a pourtant débuté en 2018. Une fois encore, nous nous rendons compte de l'impérative nécessité de mieux protéger nos concitoyens,

Français sur dix qui jugent ces appels agaçants, et neuf Français sur dix qui les trouvent trop fréquents. Si l'on dit la France divisée, voire « archipélisée », force est de constater l'unanimité du réquisitoire contre le démarchage téléphonique.

était pas un que nous en sommes réduits à devoir légiférer à nouveau sur le sujet. Si, depuis 2014, Bloctel permet aux citoyens de faire valoir leur opposition expresse à de tels démarchages, les résultats

du Sénat et de nos collègues députés, consistant à ne pas remettre en cause la philosophie du droit en vigueur afin de ne pas mettre en péril les plus de 56 000 emplois en jeu. Je crois, pour ma part, que le contexte actuel n'est pas du tout favorable à une telle remise en cause, mais nos concitoyens ne comprendraient pas que toutes

notamment de protéger les 3 millions de personnes qui ont fait la démarche de s'inscrire sur Bloctel et demandent, de façon parfaitement légitime, une vraie protection.

Nous nous félicitons des mesures visant à renforcer l'efficacité de l'et sommes d'accord avec le texte issu des travaux de la commission des lois, dont nous saluons l'effort de consensus et le travail, une fois encore de grande qualité. Nous soutenons ainsi le renforcement des sanctions en cas de manquement des professionnels du secteur, estimant que la nouvelle rédaction de l'exception contractuelle relève de cette ligne de crête qu'il convient de tenir et satisfait au pragmatisme que nous souhaitons voir prospérer

Notre groupe souhaite toutefois rétablir certaines modifications de fond introduites par l'Assemblée nationale, afin d'apporter des protections nouvelles et concrètes à nos concitoyens.

appels internationaux utilisant frauduleusement un numéro national. Nous avions déposé un amendement en ce sens ; il a malheureusement été déclaré irrecevable, mais nous conservons l'espoir qu'un compromis puisse être trouvé en CMP.

si le législateur s'est déjà attaqué au délicat sujet du démarchage téléphonique en 2014, en donnant aux consommateurs la possibilité de s'y opposer par l'inscription au service Bloctel, sous peine de lourdes sanctions administratives, force est de constater que les abus en la matière sont récurrents et confinent parfois encore au harcèlement. Depuis le début de l'examen de ce texte par le Parlement, notre rapporteur, André Reichardt, a constamment veillé à appréhender avec justesse l'enjeu central en matière de démarches téléphoniques : protéger les consommateurs sans pénaliser les acteurs économiques respectueux de la loi. Je tiens à le remercier de son travail, avant d'évoquer certains points plus précis de la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui. Ne nous y trompons pas : l'objet de ce texte est non pas d'interdire toute prospection commerciale par téléphone, mais bien de lutter contre la recrudescence de pratiques frauduleuses. À cet égard, l'interdiction générale et absolue du démarchage téléphonique aux professionnels qui vendent des équipements ou des travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d'économies d'énergie ou la production d'énergie renouvelable, prévue par les députés en seconde lecture, ne nous semble pas constituer une bonne solution. Outre qu'elle soulève un fort risque d'inconstitutionnalité au regard du principe d'égalité devant la loi et de la liberté d'entreprendre, elle pourrait s'avérer extrêmement préjudiciable pour des entreprises de ce secteur qui ne commettent pourtant aucun abus. Par ailleurs, une autre disposition du texte soulève, à mon sens, une inquiétante ambiguïté. L'article 1, à son alinéa 6, prévoit qu'un décret pris après avis du Conseil national de la consommation détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels le démarchage téléphonique est autorisé. Or la formulation employée interroge : quels types de contacts téléphoniques seraient concernés par ce cadre réglementaire ? S'agit-il de tous les appels, y compris ceux qui visent à répondre à une sollicitation expresse d'un client qui, par définition, y aurait consenti ? En raison des incertitudes suscitées par cette disposition aux conséquences non négligeables, j'ai déposé un amendement, que je défendrai tout à l'heure, visant à dissiper toute ambiguïté. Il tend à préciser que ne sont pas concernés par un tel encadrement les appels téléphoniques effectués en vue de répondre à une demande du client, avec son consentement. La crise économique inédite qui est sur le point de frapper nombre de nos entreprises impose plus que jamais au législateur de ne pas compliquer à outrance les relations commerciales respectueuses des deux parties. Pour conclure, nous saluons le travail mené sur ce texte, qui nous semblait nécessaire puisqu'il traite d'un sujet sensible tant pour nos concitoyens que pour notre tissu économique. Le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi telle qu'amendée par la commission. Merci,

est le lot quotidien de trop nombreux Français. Cet amendement, qui rejoint les analyses de plusieurs associations de protection des consommateurs, vise à reprendre le système en vigueur pour les SMS et les courriels. C'est d'ailleurs ce qui se pratique dans plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, l'Espagne et le

S'il n'a pas dit oui, alors c'est non ! Bien sûr, le modèle a ses limites, et on imagine très bien que l'accord du consommateur pourrait être obtenu au détour des conditions générales de vente ou d'utilisation, qui ne sont que trop rarement lues. À ce titre, il serait déjà plus

Bien évidemment, il y aurait toujours des clics involontaires, mais la gêne serait limitée. Il me semble surtout nécessaire, dans le cadre de la lutte conte le démarchage intrusif, de passer à une nouvelle étape en prenant le contrepied de Bloctel. Plutôt qu'un fichier de personnes ne voulant pas être dérangées, il importe de créer un fichier de citoyens ayant expressément donné leur accord pour être appelés, car c'est bien sur l'initiative du démarchage qu'il faut agir, en la laissant à la main du consommateur, et non plus de l'entreprise. La

entre 2016 et 2018, 1,3 million de réclamations émanant de 200 000 personnes ont été déposées pour les seuls inscrits au dispositif Bloctel, soit un taux de plaintes de 5

On a d'autres exemples. À la suite de la mise en place de l'au Portugal, en 2012, au Royaume-Uni, en 2018, les associations de consommateurs portugaise DECO et anglaise Which ? soulignent une baisse significative du nombre de plaintes.

pour les appels téléphoniques ? Les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités tout à fait légalement ; dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Dans cette perspective, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article, dans un souci d'harmonisation et de clarté. L'amendement

nous n'avions pas souhaité, mes chers collègues, remettre en cause la philosophie du droit en vigueur, qui repose sur un régime d'opposition expresse, l'. Même si cette décision

L'amendement n° 9 de M. Sueur tend, quant à lui, à rétablir l'article 1 A, supprimé par l'Assemblée nationale, qui prévoyait que l'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique puisse se faire par téléphone.

un centre d'appels contacte une personne vulnérable, souvent une personne âgée, et lui fait une offre ; cette personne, voulant écourter la conversation et n'ayant pas conscience de l'engagement qu'elle prend, accepte l'envoi d'un exemplaire du contrat.

De fait, instaurer une obligation d'envoi du contrat par courrier permettrait de garantir le libre choix des consommateurs et d'éviter certains abus de faiblesse, délibérés ou non.

d'un préfixe bien spécifique. Une telle disposition permettrait aux consommateurs de refuser d'être démarchés avant même d'avoir décroché et limiterait le nombre de litiges engendrés par la prospection commerciale par voie téléphonique.

Qui pourrait s'opposer à ces amendements, monsieur Sueur ? La commission, pour une raison très simple : une telle mesure pèserait uniquement sur les professionnels vertueux.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

En outre, les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019. Les relations commerciales découlant de cette pratique sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé et sont dans l'impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire totalement inexactes. Aussi, du fait de la prolifération des litiges et des mauvaises pratiques des professionnels, il convient d'interdire le démarchage téléphonique en matière de fourniture d'électricité et de gaz naturel. La parole

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

s'avère particulièrement problématique en matière d'assurances. En outre, les professionnels s'exonèrent régulièrement de leur obligation de remettre une information écrite avant toute souscription d'un contrat et n'adaptent pas les prestations proposées aux besoins des consommateurs.

M. Martin Lévrier. La rénovation énergétique des logements est une priorité pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La consommation d'énergie des bâtiments représente environ 25 % des émissions nationales les objectifs du Gouvernement en la matière sont ambitieux : une diminution de 15 % de la consommation énergétique des logements d'ici à 2023 et 500 000 rénovations performantes par an. Malheureusement, le secteur de la rénovation énergétique est particulièrement propice aux abus envers les consommateurs.

Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir adopter notre amendement ainsi sous-amendé, afin de compléter l'arsenal de la loi relative à l'énergie et au climat. Cette mesure profitera à tous : aux consommateurs, aux entreprises qui travaillent selon les règles de l'art et respectent la réglementation,

énergétique, compte tenu des nombreuses plaintes émanant de consommateurs qui font état de sollicitations intempestives, parfois agressives, et fondées sur des argumentaires commerciaux fallacieux. Nous sommes donc favorables au principe de l'interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation thermique, d'autant que celui-ci bénéficie d'une très grande visibilité, compte tenu de la politique

nous démenions pour contacter toutes celles et tous ceux qui pouvaient s'inscrire dans une démarche de rénovation efficace de leur logement- Dieu sait s'ils sont nombreux en France.

Les amendements n 31 rectifié, 13 et 21 rectifié tendent à rétablir l'interdiction de démarchage téléphonique pour les professionnels de la rénovation énergétique, de l'habitat ou de la production d'énergie renouvelable par les particuliers, que nous avons supprimée en commission. Il est patent que ce secteur est propice aux abus et aux sollicitations intempestives des consommateurs pour leur extorquer des engagements financiers en toute illégalité. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point : ces pratiques sont éminemment

Pour autant, la solution retenue par le Gouvernement et reprise dans ces amendements, soit l'interdiction pure et simple, ne nous convient pas : elle nous paraît poser un vrai problème au regard du principe d'égalité devant la loi, car tous les professionnels recourant au démarchage téléphonique pour conclure un contrat de vente sont placés dans une situation identique. En quoi les démarcheurs téléphoniques de ce secteur qui,

que les consommateurs hésitent à faire valoir leurs droits. Malheureusement, ce n'est pas en interdisant le démarchage téléphonique que ces pratiques inacceptables cesseront, la règle sera contournée par les fraudeurs, par exemple en se rendant à domicile ou en continuant d'appeler les consommateurs, alors que les professionnels de bonne foi pâtiront de cette entrave à leur liberté d'entreprendre.

ils tendent à maintenir le principe de l'interdiction générale, tout en renvoyant à un décret simple le soin de définir des exceptions en fonction de la nature de la relation contractuelle ou de la proportion d'aides publiques dans le chiffre

Le scrutin est ouvert.

Le I de cet amendement précise que la détermination des jours et horaires durant lesquels la prospection de particuliers par voie téléphonique est autorisée doit concerner toutes les sollicitations téléphoniques, qu'elles soient commerciales ou non. Il convient donc de ne pas viser seulement les sollicitations téléphoniques qui échappent aux règles d'opposition au démarchage téléphonique. En outre, n'est visé que l'encadrement, par voie réglementaire, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques sont autorisées. En effet, eu égard à la grande diversité des secteurs d'activité ainsi que des produits et services concernés, il semble très

autant. Le IV de l'amendement supprime le renvoi à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur pour désigner les professionnels réalisant des études et des sondages par voie téléphonique chargés de l'élaboration d'un code de bonnes pratiques. concernés, ce mode de désignation pose problème. Par ailleurs, eu égard à la grande diversité de nature des études et des sondages menés et des besoins auxquels ils répondent, il ne semble pas possible de déterminer la fréquence des appels, mais seulement les jours et horaires pendant lesquels les sollicitations par voie téléphonique sont autorisées. Le V du présent amendement ne prévoit que l'encadrement, par décret, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques pour la réalisation d'études et de sondages sont autorisées.

pour la réalisation d'études et de sondages lorsqu'elles sont reprises par décret. Il n'est, en effet, pas possible de sanctionner d'une amende administrative le non-respect de règles qui n'auraient pas force obligatoire. Il habilite également les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher

La séance est levée.